nous entendons, depuis quelques heures et, dans une moindre mesure, depuis quelques jours, une sorte de procès en irresponsabilité, voire en démagogie,

demandé !- Pourquoi s'efforcer d'empêcher le Gouvernement d'agir ? » D'autres ont même dit : « C'est vrai qu'à lire les apports du Sénat, on peut se demander s'ils sont utiles.

Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec le Gouvernement, il y a sans doute des divergences de vues sur la manière de faire, mais nous exerçons notre liberté, notre liberté de poser des questions. Nous voulons, dans cette période difficile, non pas vous empêcher de travailler, mais seulement assumer notre responsabilité de contrôle.

le recours aux ordonnances ou la déconcentration de la décision d'ouvrir certains commerces. Je ne vous rappellerai pas à quel point la situation est préoccupante, vous la

Les semaines qui viennent seront extrêmement sensibles et nous serons collectivement au rendez-vous. En ce qui concerne la date de sortie de l'état d'urgence sanitaire,

S'agissant du régime transitoire, qui fait l'objet d'une autre divergence entre le Gouvernement et la Haute Assemblée, je le répète : nous ne demandons pas un blanc-seing. Ce n'est pas non plus par facilité que nous proposons ce délai. Nous sommes convaincus que la sortie de l'état d'urgence sanitaire ne se fera pas du jour au lendemain. Toutes les mesures de protection de la santé des Français ne pourront s'arrêter net, sauf à maintenir l'état d'urgence sanitaire jusqu'à la disparition du dernier cas de covid-19 sur notre territoire, ce que personne ne peut considérer comme raisonnable et réaliste. L'expérience de cet été a confirmé l'utilité d'un régime pouvant prendre le relais de l'état d'urgence, faute de quoi on laisserait le virus circuler librement, ce qui est inenvisageable. Un régime transitoire, moins contraignant que l'état d'urgence sanitaire, mais permettant de protéger la santé de la population en phase de recul de l'épidémie, était déjà prévu dans le précédent projet de loi, qui n'a pu aller à son terme début octobre. La date du 1 avril 2021, retenue La date du 1 avril 2021, retenue pour ces dispositions, paraît cohérente avec la clause de caducité que le Parlement a lui-même introduite pour le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire. L'article 4 ne conduit

-de rétablir et d'adapter à l'état de la situation sanitaire actuelle, ainsi qu'aux règles de police sanitaire, les mesures d'accompagnement conçues à partir de mars dernier. Le travail du Sénat en première lecture avait prévu de circonscrire certaines habilitations ou de les inscrire directement dans le marbre de la loi. Ce n'est pas la position retenue par le Gouvernement. Compte tenu de l'évolution rapide de la situation et du renforcement des mesures de police sanitaire, il nous paraît nécessaire de disposer d'habilitations dans le but de parer à toutes les éventualités, en particulier pour répondre à la propagation de l'épidémie et à ses conséquences sur l'activité du pays. sont encore difficilement prévisibles à l'horizon des prochaines semaines. J'ajoute que cette seconde vague n'est pas identique à la précédente, et que nous devrons adapter les mesures d'accompagnement à ses spécificités dans les prochaines semaines.

hospitalier. La situation sanitaire actuelle exige des mesures clairement définies au niveau national, une territorialisation étant acceptable seulement lorsqu'elle est pertinente sur le plan sanitaire et qu'elle ne nuit pas à la compréhension des mesures. Cette lisibilité conditionne l'acceptabilité des mesures, car personne ne comprendrait que tel type de commerce soit ouvert dans tel territoire et que, quelques kilomètres plus loin, ce ne soit plus le cas. En outre, des différences territoriales risqueraient d'entraîner des brassages de populations problématiques du fait du vrai risque d'afflux de la population dans les territoires où certaines catégories de commerces resteraient ouvertes. Nous estimons qu'il est de la responsabilité du Gouvernement de définir les mesures de police sanitaire appropriées, en décidant, en tant que de besoin, de procéder à leur déconcentration.

Permettez-moi enfin de souligner que plusieurs apports du Sénat ont été conservés lors de la navette parlementaire. Je pense notamment à plusieurs précisions apportées à l'article 3 sur les systèmes d'information liés à la lutte contre l'épidémie pour permettre l'accompagnement social. propos des dispositions relatives aux infractions pénales en Polynésie française, aux règles de réunion des collectivités territoriales, à la durée maximale d'affectation dans les différentes réserves ou à la lutte contre les violences conjugales dans le cadre des mesures de confinement.

Ce virus n'épargne aucun territoire : dans l'Hexagone comme outre-mer, tous nos concitoyens sont menacés. Nous nous préparons à un choc très important dans les jours qui viennent. Nos soignants sont déjà sur le front et le pays tout entier doit être à leurs côtés. Renoncer temporairement à des libertés que nous chérissons pour sauver des vies est un sacrifice, mais c'est aussi et surtout l'honneur d'une nation qui fait de la fraternité autre chose qu'un simple principe abstrait. La parole

nous voici enfin parvenus au terme de cette discussion législative à rebondissements qui a commencé par des débats sur la prolongation du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire,

conditions regrettables si le Gouvernement doit donner le dernier mot à l'Assemblée nationale sans tenir davantage compte de notre travail. le désaccord fait partie du débat démocratique. Il peut être fécond en démocratie s'il se double de l'esprit de dialogue et si les points de vue des uns et des autres sont pris en compte.

n'a jamais marchandé l'autorisation qui lui était demandée de conférer au Gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour faire face à cette crise exceptionnelle. ses pouvoirs, en prenant soin de limiter au strict nécessaire les restrictions aux libertés individuelles et aux libertés publiques,

été en accord avec le Parlement pour que ces pouvoirs d'exception fassent l'objet d'une reconduction éventuelle par le Parlement.

la contamination de nos concitoyens par cet affreux virus ? Monsieur le secrétaire d'État, puisque nous n'avons jamais marchandé ces pouvoirs, il nous est insupportable d'entendre dire que nous ne serions pas responsables. Car, pour nous, la responsabilité ne va pas sans la vigilance et la vigilance ne va pas sans le contrôle. Comment se fait-il que ce que vous avez fait pendant sept mois, qui ne vous a donc pas paru retarder insupportablement l'action des pouvoirs publics, ne soit plus possible pour les six mois à venir ?

C'est une décision importante à prendre, les Français attendant de se préparer aux fêtes de fin d'année. Nous n'avons pas non plus refusé que l'état d'urgence se prolonge au-delà du 31 janvier ; nous avons seulement dit que, s'il devait se prolonger au-delà de cette date, il faudrait que le Parlement le vote. que le Parlement le vote. La mise en accusation du Parlement parce qu'il aurait décidé de dates butoirs au-delà desquelles les pouvoirs exceptionnels ne pourraient plus s'exercer est tout simplement une imposture dans le débat public. Ce dernier doit reposer sur des réalités

les réactions des Français dans leur diversité, joue pleinement ce rôle démocratique. Nous souhaitons que le Gouvernement ne s'isole pas au moment où c'est si difficile de faire entendre aux Français la nécessité des contraintes. Le Gouvernement, lui-même, a besoin, pour assurer l'acceptation de toutes ces contraintes, que le Parlement se prononce. Et le Parlement l'a toujours fait en vous accordant les pouvoirs que vous réclamiez ! C'est la raison pour laquelle je tiens à ce que cette mise au point soit faite. Permettez-moi d'en faire une seconde. Monsieur le secrétaire d'État, vous le savez certainement,

Ce n'est pas parce que vous ne faites plus le confinement et le couvre-feu que vous n'avez plus besoin de recourir aux moyens de l'état d'urgence sanitaire, qui sont les mêmes que ceux du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Cette invention du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire ne répond qu'à une exigence psychologique, certainement pas juridique. Dans le cadre

en mode mineur, au régime de l'état d'urgence, qui prévoit tout à fait, parmi les neuf catégories de dispositions restrictives pour les libertés susceptibles d'être prises, celles dont vous aurez besoin. Elles sont, d'ailleurs, exactement les mêmes que celles auxquelles vous avez eu recours dans le cadre de la loi du 9 juillet. superposé inutilement deux régimes. Nous vous l'avons dit dès le 9 juillet ; ne recommencez pas ! Nous sommes d'accord sur la nécessité de ne pas sortir d'un seul coup du régime des contraintes qui existent et sur la nécessité d'une transition. Vous voyez, monsieur le secrétaire d'État, je viens vers vous ; vous pourriez faire l'effort de venir vers nous aussi. Et je vous remercie d'être attentif à ce que je vous dis S'agissant de l'ouverture de certains commerces, où avez-vous vu que nous voulions procéder par catégorie, par territoire, par des mesures d'ordre général, prendre le risque, selon vos de « brassage de populations » qui seraient attirées par la différence de régime d'un territoire à l'autre ? Là encore, nous vous donnons les moyens d'apprécier les situations

Cela me paraît tout à fait simple à organiser. Ce n'est pas seulement moi qui ne comprends pas ; ce sont aussi des millions de Français qui voient chaque jour vingt millions de personnes rejoindre leur travail, qui voient chaque jour douze millions d'enfants rejoindre l'école, un million de professeurs assurer l'enseignement dans les écoles, qui se demandent pourquoi le commerce de chaussures de Villedieu-les-Poêles doit être fermé et pour quelle raison son ouverture constituerait un danger pour la sécurité sanitaire. Du bon sens, Du bon sens, du respect pour le Parlement, une capacité de comprendre que, quand on agit seul, on est plus faible que quand on agit en accord avec le Parlement

n'en est pas une puisqu'il s'agit du texte initial que nous avons examiné la semaine dernière. Nous l'avons amendé en vain puisque consigne a été donnée aux députés de La République En Marche de rétablir le texte initial sans tenir compte ni des apports du Sénat ni des avis divergents au sein même de son hémicycle. hémicycle. Quelle pitoyable image du Parlement est renvoyée à nos concitoyens qui, plus que jamais, font preuve d'une certaine abnégation face aux mesures de restriction de libertés qui leur sont imposées

ne lui soit pas acquis et que sa position redonne du sens à notre démocratie et au rôle fondamental de la représentation nationale. Aujourd'hui, à l'heure où les libertés publiques sont restreintes, le dernier lieu de débat démocratique devrait être hissé au plus haut rang par l'exécutif. Or c'est c'est au sommet d'un petit cercle de réflexion autour du Président de la République, qui ne se cantonne même plus au Conseil des ministres, mais à un conseil de défense dévié de sa nature première, que les décisions se prennent. Qu'en est-il vraiment, monsieur le secrétaire Jean-Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, disait il y a peu qu'« il y a un risque d'accoutumance aux mesures de contrôle. Dans certains cas, les pouvoirs publics peuvent se dire que, après tout, si une mesure n'a pas entraîné de levée de boucliers, on continue

à organiser ! Cette deuxième vague était plus que prévisible, mais vous feignez aujourd'hui la surprise, car votre priorité est de sauver la face d'un système qui est arrivé en bout de course. Il est aisé de brandir les pseudo-menaces contre les grandes plateformes numériques qui seraient les ennemies de l'État, alors qu'elles étaient jusque-là parfaitement imbriquées- imbriquées- elles le sont d'ailleurs toujours, derrière les faux-semblants -dans le système libéral et capitaliste que vous prônez. Il est également aisé de s'emporter dans de grands plaidoyers en faveur de nos soignants, qui n'ont pas attendu la covid-19 et ses vagues successives pour tirer la sonnette d'alarme d'un hôpital public exsangue. Nous étions avec eux hier comme nous le sommes aujourd'hui. Mes chers collègues, nous vous proposerons de nouveau, par voie d'amendement, de retenir la date du 14 décembre prochain comme fin du régime d'état d'urgence sanitaire pour affirmer, comme nos collègues députés, que nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement ; que nos voix comptent tout autant ; que le pouvoir législatif n'est pas le bras armé d'un exécutif retranché sur son conseil de défense pour faire la pluie et le beau temps dans la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour les six mois qui viennent. Ces préoccupations sont fondamentales pour notre démocratie, quelles que soient les circonstances. Dans le même sens, nous vous demanderons de nouveau de mettre en place un comité de suivi national de la crise, véritable comité de santé publique permettant un contrôle démocratique efficient et une réelle participation de toutes et de tous aux décisions. La balance entre taux de mortalité et équilibre économique n'a que trop tangué entre les mains de l'exécutif. Il est de notre devoir d'apporter notre lecture de la crise sanitaire en cours le plus sérieusement et le plus régulièrement possible. Aussi, comme en première lecture, nous nous opposerons à la philosophie globale de ce texte, que la majorité sénatoriale n'a malgré tout pas remise en cause

nous vous annoncions la tempête en soulignant votre manque de concertation. Ces propos ne s'adressent pas à vous personnellement : nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises et certains de vos collègues devraient s'inspirer de votre capacité d'écoute

Comme je le disais à votre collègue Mme Bourguignon il y a une semaine, pour être unis, il faut la volonté des deux parties. Nous vous annoncions la tempête en vous parlant des commerçants, seuls Français à qui l'on interdit de travailler. Tout le monde peut aller à l'école, au travail, dans le métro, mais pas chez le coiffeur, même pas chez le libraire. Nous vous annoncions la tempête en vous signalant

Au-delà des commerçants, que vous entendez aider, je pense à tous les métiers de l'événementiel, du serveur au loueur de tentes, en passant par les artistes. Combien se retrouvent dans un marasme tel que le dépôt de bilan risque d'être leur seule issue ?

Il est vrai- je l'ai déjà dit -que l'on ne forme pas une infirmière en deux mois et que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe à l'hôpital. Mais avouez que, si vous aviez trouvé l'« argent magique » plus tôt, si vous l'aviez consacré au système de soins dès 2017, nous n'en serions pas à déprogrammer des opérations,

J'ai bien entendu notre ministre de la santé piquer une grosse colère à l'Assemblée nationale et citer une série d'exemples pour provoquer l'émotion. Il a raison : toute vie mérite d'être vécue et doit être sauvée quoi qu'il en coûte. Mais on ne dirige pas à coups d'émotions.

lorsqu'on vous parle de la dépression des Français et de la faillite de leurs entreprises ? La pauvreté n'aura-t-elle pas un impact sur les familles, sur les enfants ? Cette fois-ci, c'est bien à vous que je pose la question La culpabilisation des sénateurs, qui, au motif qu'ils demandent à exercer pleinement leur mission constitutionnelle de contrôle de l'action du Gouvernement, n'auraient pas conscience de la gravité de la situation, n'est pas acceptable.

Quand on voit la qualité du travail de notre rapporteur, notamment son examen rigoureux des demandes d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance ; quand on voit, parallèlement, la facilité avec laquelle les députés renoncent à leur mission de législateur, on ne peut pas porter de telles accusations. Certes, vous avez à résoudre la quadrature du cercle ... Eh oui ! Votre rôle n'est pas simple. Il l'est d'autant moins que vous vous entêtez à agir seuls et, surtout, à ne rien retenir de ce que l'on peut vous proposer. Nous vous demandons de rouvrir les librairies et vous interdisez les ventes de livres autrement que par internet. Nous vous demandons de laisser les préfets juges ce que l'on peut faire en fonction des situations sanitaires inégales que connaît notre territoire et vous nous répondez : « On ne revient pas sur la parole du Président de la République ! » Nous vous demandons d'associer le Parlement aux décisions

des nuances, des différences ou des désaccords reviendrait à priver le Gouvernement de toute possibilité d'action face à cette crise. Or c'est inexact ! M. le rapporteur l'a rappelé à l'instant : jamais le Parlement n'a hésité à donner tous les pouvoirs nécessaires au Gouvernement pour lutter contre l'épidémie. D'ailleurs- peut-être ne l'avez-vous pas noté

l'état d'urgence et définir ses modalités. Ce n'est pas faire injure au Gouvernement que de dire qu'il est en grande difficulté dans ses relations avec nos concitoyens ; que la politique appliquée aujourd'hui pour lutter contre l'épidémie n'est pas comprise,

Des dizaines de milliers de nos concitoyens ont été touchés par la covid ou le sont encore ; 38 000 d'entre eux sont morts et le nombre des décès continue de progresser, rappelant tristement les chiffres d'avril

tout doit être mis en oeuvre dans les prochains mois pour améliorer rapidement la situation sanitaire, limiter le nombre de décès et sortir au plus vite du confinement. Nous sommes tous conscients qu'il faut donner à l'exécutif les marges de manoeuvre dont il a besoin pour agir dans cette situation critique. Pour autant, ces réponses ne doivent pas avoir pour postulat l'affaiblissement du Parlement. Parlement. Pour permettre au Gouvernement de déroger aux règles de droit commun, le vote d'une loi est essentiel. À cet égard, l'exécutif doit satisfaire un certain nombre de demandes : il importe que le Gouvernement procède régulièrement à une évaluation de la situation,

éventuelle. À mon sens, l'instauration d'un régime d'exception qui contraint les libertés de nos concitoyens exige un débat démocratique régulier. Il s'agit là d'un gage d'acceptation des mesures envisagées. En contournant le débat, on ne fera que renforcer la défiance des Français. Le succès de ces mesures dépend de la participation active et de l'adhésion de tous. Il faut le rappeler. Par ailleurs, je me félicite tout particulièrement que le Sénat ait adopté, à l'unanimité, un amendement présenté par M. le rapporteur : il s'agit de permettre au préfet d'autoriser, à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires

Dans ces temps difficiles, une concertation étroite avec les collectivités territoriales et les corps intermédiaires serait de nature à conforter la légitimité des politiques publiques et, partant, de l'exécutif. Nos institutions ne doivent pas fonctionner en mode dégradé.

Pour lui, c'est le travail qui serait leur quotidien : comme si nous, parlementaires irresponsables, passions notre temps à chercher des noises au Gouvernement, tandis que les soignants se battent pour sauver des vies Monsieur le secrétaire d'État, nous nous inclinons toutes et tous devant le travail de nos soignants et nous savons tout ce que nous leur devons. Mais sachez aussi qu'il y a ici des parlementaires, des collaborateurs, des fonctionnaires et, autour de nous, des membres de nos familles atteints de la covid-19. Sachez que certains d'entre nous sont passés à deux doigts du pire. Votre tâche est certes difficile, mais la maladie que nous avons vécue dans notre chair nous autorise, me semble-t-il, à ne pas tout accepter d'un gouvernement pratiquant une verticalité de plus en plus pesante. Vous nous proposez de vous dispenser du débat parlementaire jusqu'en février 2021. On ne décrète pas l'union nationale de manière autoritaire, en réduisant le Parlement au silence. Sur le sujet si grave de la pandémie, l'unique recours aux ordonnances, pendant un temps si long, est inacceptable ! Nos institutions démocratiques sont déjà éprouvées par la multiplication des états d'urgence. Le risque d'accoutumance aux régimes exceptionnels

Déjà fragilisés par le premier confinement, nos petits commerces subissent la concurrence déloyale de la vente en ligne. Leur ouverture pourrait cependant être assurée, comme en Belgique, dans le strict respect des protocoles sanitaires et sous le contrôle du préfet et des maires. Les incohérences récurrentes qui frappent les décisions du Gouvernement ont même eu pour effet de provoquer la colère d'élus locaux de tous bords ; certains d'entre eux ont ainsi pris des arrêtés illégaux pour les contrer. J'ajoute que votre soutien reste gravement lacunaire pour toute une frange de la population tombée dans la grande précarité, notamment nos jeunes. nos jeunes. Pourquoi ne pas élargir les conditions d'octroi du RSA aux personnes sans ressources âgées de 18 à 25 ans ? Face à l'urgence de la situation, cette proposition devrait déjà être à l'étude. Depuis le début de l'épidémie, députés et sénateurs sont pleinement mobilisés et demandent une gestion collégiale de la crise. Puisque vous restez sourds à cette requête, les élus du groupe Écologiste- Solidarité et Territoires voteront contre ce projet de loi ! La parole

je pourrais décliner, comme en première lecture, le triste état des lieux de la situation sanitaire, partagé par nos voisins européens, ou amorcer une approche comparative sur les moyens de droit pris pour y répondre. Les dernières données sur la situation sanitaire en France semblent, ce soir, parler d'elles-mêmes. Ces chiffres sont inquiétants, car nous savons qu'ils ne pourront s'améliorer à très court terme. Ils sont préoccupants, aussi, car en découlent des enjeux éthiques d'une importance cardinale. Je pense aux choix que seraient amenés à faire les soignants dans le cas où ils ne seraient pas en mesure d'apporter des soins à chacun, ou encore aux patients

à une quelconque irresponsabilité des autres. Mais il me semblait important, pour ouvrir mon propos, de rappeler d'où nous parlons ce soir. Aucune décision n'est prise de gaieté de coeur, avec arrière-pensée ou sans une responsabilité bien pesée. Je salue d'ailleurs le choix fait par notre rapporteur de consentir à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Sur ce point, et à rebours de l'opposition manifeste qui peut ressortir du rapport, les positions n'apparaissaient pas, sur le fond, irréconciliables au commencement. Une durée de deux semaines sépare les échéances adoptées par les deux chambres. De même, prolonger le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1 avril 2021 ne revient pas, à notre sens, à donner un blanc-seing au Gouvernement pour cinq mois ni à nous dessaisir de nos pouvoirs. D'une part, une autre échéance, celle de l'état d'urgence sanitaire lui-même, interviendra entre-temps, et le Parlement pourra alors, seul, autoriser la prolongation de ce régime. D'autre part, le régime transitoire précité confère au Gouvernement des outils- une faculté -qu'il pourrait mettre en oeuvre si, et seulement si la situation l'exigeait, ce sous le contrôle du juge, qui peut statuer en référé, mais aussi sous le contrôle renforcé du Parlement. La prolongation de l'autorisation de mise en oeuvre des systèmes d'information de santé jusqu'au 1 avril 2021, en ce qu'elle assoit la stratégie « tester, tracer, isoler », nous semblait également importante, incompatible avec la position que notre assemblée avait pu adopter au mois de mai sur un précédent texte d'urgence, lorsqu'elle avait consenti, avec l'Assemblée nationale, à fixer le terme de l'utilisation de ces systèmes à six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, tel que déclaré en mars. Enfin, nous nous accordons sur ces travées sur la nécessité de prolonger ou de réactiver un certain nombre de mesures d'urgence économique et sociale. Je pense, notamment, au dispositif d'activité partielle ou au fonds de solidarité. Notre Notre divergence réside donc dans la méthode : il n'est pas aisé de concéder des habilitations, mais les habilitations prévues par le Gouvernement visaient, pour la totalité d'entre elles ou presque, des dispositions déjà prises sur le fondement de précédents textes. Ces mesures ont une ambition cardinale : protéger les plus fragiles dans la période que nous vivons. Le défi est similaire à la situation des commerces non alimentaires de proximité. Depuis l'examen du texte en première lecture, des mesures indispensables ont été annoncées pour répondre aux difficultés. Il ne s'agit en aucun cas d'opposer ce qui participerait de l'essence de notre action à ce qui n'en constituerait qu'un agrément ni, plus généralement, d'opposer la protection de la vie à l'économie.

Parallèlement, le nombre de contaminations continue d'augmenter, tout comme celui du nombre d'admissions de malades à l'hôpital et dans les services de réanimation. Devant ce constat, la représentation nationale doit tenir son rôle : celui de se montrer responsable face à l'épidémie et d'agir pour la maîtriser. Aussi, le groupe du RDSE et moi-même ne discutons pas l'importance qu'il y a à proroger l'état d'urgence sanitaire- nous l'avons déjà exprimé. Si nous sommes généralement opposés à être dépossédés de notre mission, aujourd'hui la raison et l'urgence de la situation l'emportent sur les principes. Toutefois, nous regrettons que nos collègues députés n'aient pas retenu les initiatives mesurées du Sénat en faveur du maintien d'un contrôle parlementaire tout au long de l'état d'urgence sanitaire.

Naturellement, nous avons conscience de la difficulté et de l'ampleur de la tâche. C'était encore plus vrai au mois de mars dernier ... À ce propos, quelles leçons avons-nous tirées depuis Aujourd'hui, à peine la règle pensée, chacun lui cherche des exceptions et des dérogations. Les débats se multiplient et diffusent le doute et l'inquiétude, tant parmi les élus que parmi nos concitoyens. Il faut rechercher la cohérence, il faut clarifier les dispositifs et ne pas laisser la moindre place au flottement et à l'indécision, qui alimentent un sentiment d'arbitraire et d'illégitimité de la décision. Ces remarques très générales valent aussi bien pour l'ouverture des commerces que pour la gestion des écoles ou l'organisation des élections. Cela a été dit, le Sénat avait unanimement voté en faveur de la possibilité d'adaptations locales par le préfet afin d'autoriser l'ouverture des commerces de vente au détail. Nous avions entendu et relayé la détresse des maires, qui n'étaient pas, contrairement à ce qui a été déclaré, irresponsables. Ils étaient seulement inquiets, face aux situations dramatiques émaillant les territoires. L'Assemblée nationale n'a pas souhaité s'accorder avec cette disposition. Nous le regrettons. Nous espérons que les principes et les règles s'appliqueront de manière pérenne et ne créeront pas d'iniquité et de concurrence déloyale. Les enjeux sont les mêmes s'agissant des élections locales à venir. Faudra-t-il les repousser, et à quelle date ? Si cette solution devait être envisagée, le report permanent ne pourrait être la seule réponse. Là aussi, il ne faudra pas se borner à repousser le problème, sans mettre à profit les prochains mois pour imaginer des outils de substitution conformes à nos règles démocratiques. Enfin, je voudrais terminer par un point, certainement le plus important. Partout dans notre pays, la misère sociale augmente de façon préoccupante, mettant un trop grand nombre de nos concitoyens dans une précarité financière et humaine. La pauvreté s'accentue, nourrie par les défaillances en cascade d'entreprises et touchant en premier lieu les plus vulnérables d'entre nous. Elle frappe encore plus ceux qui étaient déjà trop souvent laissés en marge de notre société, ceux qui souffrent plus que d'autres de l'isolement ou de la précarité de l'emploi. Sans minimiser tous les dispositifs déjà mis en place pour le soutien à l'économie de notre pays, il est urgent que le Gouvernement apporte aussi des réponses et des solutions concrètes pour qu'aucun de nos concitoyens ne soit laissé sur le bord du chemin. Pour conclure, le groupe du RDSE est pleinement satisfait que notre assemblée ait fait le choix de réexaminer le texte- une fois n'est pas coutume ! Nous nous associerons par un vote favorable à cette nouvelle lecture, qui nous semble apporter des garanties sur le rôle essentiel du Parlement dans la gestion de cette crise.

J'entends à la fois l'enthousiasme et l'absence de surprise face à ces propos ... Je m'en doutais un peu ! L'avantage que me confère ma position de dernier orateur est de ne pas avoir besoin de développer très longuement les motifs pour lesquels le groupe Les Républicains votera ce texte. mes chers collègues, le Gouvernement nous demande, face à la situation sanitaire du pays, de l'autoriser à faire usage de l'état d'urgence pour une durée